au risque de nuire au suspense, j'indique d'emblée que la commission des finances vous recommande d'adopter les 2,5 milliards d'euros de crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». Cette recommandation ne s'en accompagne pas moins d'un sentiment mitigé suscité par un projet de budget dont les équilibres sont critiquables sur des points cruciaux. J'en mentionnerai quelques-uns. Première observation : l'effort financier au bénéfice des anciens combattants tend à se déformer dans le sens d'une accentuation de la part des avantages sélectifs aux dépens des prestations à caractère universel. Cette évolution pose un problème d'équité. Elle résulte notamment des dépenses fiscales. Celles-ci pèsent 751 millions d'euros, soit 31 % des crédits de la mission, et devraient s'alourdir mécaniquement compte tenu de la perspective d'une augmentation

cette accentuation de la sélectivité s'accompagne d'une sous-indexation chronique des interventions financées par la mission, qui renforce l'acuité des interrogations sur la distribution des transferts qu'elle met en oeuvre. Le nombre des anciens combattants baisse, de l'ordre de 5 % par an. Les crédits de transferts crédits de transferts baissent de 3,1 %, soit un peu moins, mais ce décalage n'est dû qu'à l'extension en année pleine de revalorisations acquises les deux années précédentes. Il faut encore noter l'impact des deux mesures nouvelles formalisées dans les articles rattachés. avec 6,5 millions d'euros, elles ne présentent pas les mêmes enjeux que le choix de ne pas indexer les différentes prestations, qui dégage une économie de plus de 23 millions d'euros. Ma troisième observation se déduit de la précédente : le projet de budget adresse un signal négatif aux anciens combattants, celui d'une perte régulière de pouvoir d'achat des prestations qui leur sont adressées et, avec elle, celui d'une dévalorisation de la reconnaissance de la Nation envers envers eux. Le projet de loi de programmation des finances publiques et sa traduction triennale pour les anciens combattants prolongent cette inquiétude légitime. Il faut rapidement corriger cette impression. Dans ces conditions, et c'est ma quatrième observation,

de l'établissement, opérateur de l'État, qui conduit une restructuration à encourager ne compensent pas tout, mais il faut plutôt s'en féliciter. L'engagement de la transformation de l'Institution nationale des Invalides, l'INI, opérateur de l'État, est également un motif de satisfaction. Ma cinquième observation me conduit à m'interroger sur les moyens de mieux agencer notre politique de reconnaissance envers les anciens combattants. Outre la préoccupation essentielle de ne pas leur imposer une part disproportionnée dans la contribution au rétablissement de nos comptes publics, je crois qu'il conviendrait de réfléchir à l'adéquation entre notre appareil de reconnaissance et la nouvelle sociologie des combattants. La quatrième génération du feu présente en effet des particularités qu'il faudrait mieux prendre en compte. De la même manière, certaines situations individuelles devraient faire l'objet d'améliorations. Il en va ainsi de celle des forces qui protègent notre territoire contre les actions terroristes dans le cadre de l'opération Sentinelle ou encore des aidants des très grands invalides de guerre.

ma présentation en relevant, par une dernière observation, que le projet de budget pour 2018, mais également la mission telle qu'elle est programmée pour les années 2018 à 2020 me semblent faire l'impasse sur des éléments importants. Le service universel obligatoire d'un mois qui pourrait remplacer la Journée défense et citoyenneté n'est pas budgété dans la loi de programmation des finances publiques. Je rappelle que la JDC, qui dure un jour, coûte environ 150 millions d'euros au budget de l'État. La réorientation des missions de réparation des spoliations antisémites financées par le programme 158 vers une politique plus proactive consistant à identifier des oeuvres spoliées et les ayants droit des réparations afin de lever les parts réservées des indemnisations ne fait l'objet d'aucune traduction dans traduction dans le projet de budget et pas davantage dans le projet de loi de programmation pluriannuelle. Moyennant ces observations en guise d'avertissement, je vous confirme la décision de la commission des finances d'adopter les crédits de la mission. La France a combattu et la France combat. Elle fait son devoir. Le devoir de tous les Français est de marquer leur reconnaissance envers ses anciens combattants, les jeunes et les moins jeunes. Nous veillerons attentivement à ce qu'il en soit mieux ainsi dans les prochaines lois de finances. La parole est à M.

Les propos que je vais tenir sont donc les siens, madame la secrétaire d'État. La commission des affaires sociales a émis, la semaine dernière, un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Pour autant, même si elle a apprécié les échanges qu'elle a pu avoir avec vous, madame la secrétaire d'État, elle ne peut se satisfaire d'enregistrer purement et simplement le lien mécanique entre le déclin démographique des anciens combattants et le recul du budget. Chaque année, nous constatons que les anciens combattants de la guerre d'Algérie vieillissent, tandis que les jeunes anciens des opérations extérieures, les OPEX, restent peu nombreux. En 2018, les effectifs des anciens combattants diminuent de près de 5 % et les crédits de la mission, de 3 %. Nous pensons qu'une partie de la substantielle économie réalisée, qui s'élève à 76 millions d'euros, aurait pu être mise à profit pour corriger certaines des iniquités qui persistent dans l'application du droit à réparation. Bruno Gilles en a identifié deux dans son rapport, liées à la guerre d'Algérie. Il y a, tout d'abord, la question de l'attribution de la carte du combattant pour quatre mois de service en Algérie entre juillet 1962 et juillet 1964. Alors que 627 d'entre eux y ont été reconnus « morts pour la France », comment est-il possible de refuser la qualité de combattant aux hommes qui ont servi durant cette période ? Il n'est pas ici question d'ouvrir un débat historique sur la guerre d'Algérie ou de venir perturber les relations entre nos deux pays. Au contraire, il faut plutôt considérer qu'il s'agissait là d'une opération extérieure. Le coût de cette mesure serait de l'ordre de 18 millions d'euros par an ; elle pourrait donc être financée dans le projet de loi de finances pour 2019. Il convient aussi de mettre un terme à l'injustice dont sont victimes les anciens supplétifs de statut civil de droit commun, ces pieds-noirs qui ont servi dans les harkas et les autres formations supplétives sans que leur engagement soit reconnu jusqu'à ce jour. Ainsi, le législateur leur a toujours refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance. Une décision du Conseil constitutionnel leur avait pourtant temporairement donné satisfaction, mais l'administration n'a pas accédé à leurs demandes. Environ 70 personnes seraient concernées, ce qui représente un coût, minime, de 260 000 euros par an. Il faut agir dès cette année, madame la secrétaire d'État, en faveur de ces femmes et de ces hommes, qui vivent souvent dans une situation précaire. C'est l'objet

dans la suite de nos débats. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

je souhaite aujourd'hui porter la voix des associations représentatives du monde combattant, qui ont toute ma considération et dont j'ai eu plaisir à auditionner les représentants locaux, ces dernières semaines, dans mon département, le Calvados. Je débuterai mon intervention en soulignant combien ces associations regrettent l'absence d'un secrétariat d'État chargé spécifiquement des anciens combattants et de la mémoire au sein de l'actuel gouvernement. Le monde associatif représentatif des anciens combattants et des victimes de guerre s'inquiète d'une telle absence. Ces associations estiment très justement que, moralement et symboliquement, les anciens combattants sont un facteur essentiel, aussi bien pour la transmission de la mémoire que pour le bon déroulement des cérémonies patriotiques. Elles estiment également que, pour l'opinion publique, il eût été indispensable que la liste des membres du Gouvernement fasse état, clairement et lisiblement, de leur existence à travers l'affectation d'une personne dédiée à cette fonction spécifique. Indispensable aussi pour le devoir de mémoire, afin mémoire, afin que certains événements historiques tragiques ne se reproduisent plus ; mémoire pour toutes ces victimes, tous ces soldats morts ou blessés pour la France. Jamais les citoyens français ne doivent oublier les sacrifices consentis par leurs aînés hier et par leurs pairs aujourd'hui pour assurer notre droit à vivre libres, égaux et dans la fraternité. Ce budget 2018 des anciens combattants, de la mémoire et du lien armée-Nation au travers de la jeunesse s'établit à 2,46 milliards d'euros, en baisse de 3 % par rapport à 2017. Chaque année, le ministère justifie ces reculs par la diminution du nombre d'anciens combattants. Je note, surtout, que ces réductions budgétaires aboutissent à ce que les différentes générations du feu ne soient toujours pas traitées de la même manière. Bien sûr, le groupe socialiste et républicain a parfaitement conscience qu'il n'est, hélas, pas possible, dans un contexte budgétaire contraint, de remédier à court terme à toutes les inégalités que subissent nos concitoyens. Néanmoins, nous tenons à souligner que les injustices dont nous débattons aujourd'hui pénalisent depuis des années, voire des décennies, ceux qui, ayant consacré leur vie à la Nation, méritent pourtant des réponses claires. Nous regrettons tout particulièrement que la hausse du point de retraite, confirmée pour septembre dernier- et qui était une décision du Gouvernement précédent -ne soit pas pérennisée,

au-delà de la baisse des effectifs des bénéficiaires des crédits discutés aujourd'hui, l'extension, par exemple, depuis le 1 octobre 2015, des critères d'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à une OPEX pendant au moins 120 jours va nécessairement engendrer une augmentation légitime du budget, particulièrement quand ces bénéficiaires arriveront à l'âge de la retraite. Rien, dans ce budget, ne semble anticiper cette évolution, ce qui confirme notre crainte d'un effet de ciseaux entre l'entrée de ces nouveaux bénéficiaires et la baisse continue du budget des anciens combattants, obérant la capacité des gouvernements successifs à faire des propositions nouvelles, voire à tenir des engagements pris. De même, certains sujets auraient mérité de trouver une issue favorable en cette année 2018. Je pense en particulier à l'attribution de la carte du combattant à ceux qui, ayant séjourné en Algérie entre juillet 1962 et 1964, attendent depuis cinquante ans d'être enfin reconnus par la Nation. Je citerai également le droit à l'indemnisation pour les pupilles de la Nation dont les parents ont été reconnus

encore l'extension de la campagne double, à attribuer en fonction du temps passé sur un théâtre de guerre et non plus en fonction des actions de guerre, ou encore l'assouplissement du dispositif de la demi-part fiscale supplémentaire, de façon à en faire bénéficier toutes les veuves d'anciens combattants, quel que soit l'âge du décès du conjoint. J'ai été particulièrement alertée par la situation financière de nombreuses veuves, qui subissent une chute de revenus importante après le décès de leur mari, au point, pour certaines d'entre elles, de se retrouver dans un extrême dénuement. Cela n'est pas acceptable. Je souhaite aussi me faire l'écho des inquiétudes qui s'expriment à propos du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui se veut constant alors que ses missions s'élargissent et qu'un grand nombre d'anciens combattants ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté. L'ONAC-VG doit aujourd'hui accompagner des publics nouveaux, aux demandes plus importantes. De même, si l'Office poursuit sa modernisation, celle-ci doit se faire en préservant les indispensables liens de proximité tissés avec les bénéficiaires et les associations locales représentatives du monde combattant. 2018 devrait être une année de réflexion sur l'évolution stratégique de l'ONAC-VG qui préparera le contrat d'objectifs et de performance entrant en vigueur en 2019. Il nous paraît essentiel de consolider le réseau territorial actuel. Autrement dit, malgré l'émergence de grandes régions, tout doit être fait, dans les années à venir, pour conserver le maillage départemental de l'ONAC-VG et mieux harmoniser les pratiques entre territoires. Alors, bien sûr, il y a aussi des points positifs dans ce budget. Je note, en lien avec le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la hausse de près de 25 % des moyens dédiés à la politique de mémoire 8 millions d'euros seront versés à la mission du centenaire et plus de 10 millions d'euros seront consacrés à l'entretien et à la rénovation des sépultures, et ce en lien avec le projet d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité des sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre. Je pense également aux articles 50 et 51 du projet de loi de finances, rattachés à cette mission. Le premier prévoit une revalorisation de 100 euros de l'allocation de reconnaissance versée aux harkis, ainsi que de l'allocation viagère en faveur de leurs conjoints survivants. À cela s'ajoute, avec l'article 51, une mesure d'équité permettant le calcul des pensions d'invalidité et des pensions de réversion antérieures à 1962 au taux du grade, et non plus au taux forfaitaire du soldat. Avec ces deux articles rattachés, les choses vont dans le bon sens, mais doivent toutefois être relativisées au regard du faible nombre de personnes concernées. Loin de toute polémique, ce qui ne serait pas à la hauteur du monde combattant, et malgré quelques regrets et réserves, madame la secrétaire d'État, les sénateurs du groupe socialiste et républicain prendront leurs responsabilités, voteront les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », afin de soutenir les quelques avancées de ce budget

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au coeur des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale, je rends ici hommage à nos militaires vétérans et à leurs familles pour les sacrifices consentis à la défense de la France, sur son sol et ailleurs. La patrie se doit de leur montrer sa reconnaissance. Dans cette optique, je salue la décision du Gouvernement de stabiliser les crédits et les emplois de cette mission, la diminution de l'ordre de 3 % des crédits s'expliquant en partie par la baisse naturelle du nombre de bénéficiaires des différents dispositifs. Le programme 167 est en hausse de 4,5 millions d'euros. La croissance importante du budget en faveur de la mémoire pour l'année 2018 est une nécessité pour faire du centenaire de la Grande Guerre un événement de rassemblement national et de souvenir collectif majeur. La fin du cycle des commémorations de 14-18 doit être l'occasion de remettre au centre de notre politique la transmission à notre jeunesse d'une pédagogie renouvelée sur notre politique de défense, et c'est ce qui apparaît dans ce budget. Le programme 169 est, quant à lui, en baisse de 80,6 millions d'euros. Cette tendance est confirmée par le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022. La décroissance naturelle du nombre de bénéficiaires ne prend pas en compte des mesures qui auront une incidence budgétaire à moyen terme, comme l'extension, depuis le 1 octobre 2015, des critères d'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à une OPEX pendant au moins 120 jours. Alors, que retenir principalement de ce budget ? L'augmentation de deux points de la retraite du combattant représente un effort qui était nécessaire. Le budget de l'action sociale de l'ONAC-VG, maintenu à 26,4 millions d'euros, permettra de soutenir les anciens combattants, conjoints survivants, la quatrième génération du feu et les victimes d'actes de terrorisme. Nous nous réjouissons également de l'investissement sur cinq ans de 50 millions d'euros de rénovation des bâtiments de l'Institution Nous saluons les initiatives concernant l'entretien et la valorisation des monuments et hauts lieux de la mémoire nationale et le tourisme mémoriel. Nous approuvons les mesures prises pour corriger des inégalités connues de longue date, comme la revalorisation de 100 euros de l'allocation de reconnaissance versée aux harkis et l'alignement des pensions militaires d'invalidité. Malgré ces mesures attendues et justes, quelques interrogations demeurent. Je pense notamment à la carte « 62-64 » qui n'est toujours pas accordée aux anciens combattants d'Algérie restés après les accords d'Évian. Qu'attendons-nous pour réparer cette injustice ? encore à la révision de l'indemnisation des pupilles de la Nation dont les parents sont morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, ou bien à la revalorisation de la pension de base des conjoints survivants des grands invalides de guerre. Je pense également à la situation des supplétifs de statut civil de droit commun. Il est regrettable que certains aient vu leurs droits reconnus en justice quand d'autres ont été déboutés pour des questions de forme. Il s'agit de mettre fin à une rupture d'égalité qui a d'ailleurs été dénoncée par le Conseil constitutionnel et qui ne devrait pas avoir d'incidence financière importante au regard du nombre peu élevé de personnes concernées, Ce budget, madame la secrétaire d'État, est satisfaisant malgré la baisse des crédits. Il conforte les dispositifs de reconnaissance et de réparation, et corrige plusieurs inégalités, même si certaines demeurent. Il accompagne, par des crédits supplémentaires, le cycle du centenaire et la modernisation des opérateurs du monde combattant, et ce dans un contexte de réduction du déficit public, nous en sommes tous conscients. Nous prenons acte des efforts engagés et espérons que d'autres avancées nécessaires, dont celles que je viens d'évoquer, verront le jour au cours de la législature, pour le respect, la dignité et la reconnaissance que nous devons aux combattants et à leurs familles. Tous ces éléments vont dans le bon sens et, pour cela, madame la secrétaire d'État, mon groupe votera ces crédits. Néanmoins, dans cette mission plus que dans toute autre, il s'agit, au fond, de réfléchir à ce qui fait de nous une Nation, aux valeurs qui justifient le combat, les blessures, le sacrifice ultime de nos soldats. Comme le disait très justement Simone Veil : « Je n'aime pas l'expression de devoir de mémoire. Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. »

messieurs les présidents de commission, monsieur le rapporteur spécial, cher Marc, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le budget 2018 de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Le budget total de cette mission, pour 2018, s'élève à 2,46 milliards d'euros. Ce budget, vous le savez, traduit la reconnaissance et la solidarité de la Nation à l'égard des anciens combattants. Il témoigne non seulement de l'hommage rendu par la Nation à ceux qui lui ont sacrifié une part d'eux-mêmes, mais aussi de la volonté de l'État de transmettre la mémoire de notre histoire et d'affermir les liens entre la Nation et son armée. Ce budget préserve et consolide intégralement les droits des anciens combattants, dans la mesure où l'ensemble des dispositifs budgétaires et fiscaux est maintenu. Ce budget comprend deux mesures nouvelles, qui répondent à des impératifs d'équité et d'amélioration des dispositifs en vigueur : l'article 50, tout d'abord, qui prévoit une revalorisation de 100 euros de l'allocation de reconnaissance et de la rente viagère versées aux anciens membres des formations supplétives ; l'article 51, ensuite, qui instaure, à compter du 1 janvier 2018, un alignement des pensions militaires au taux du grade, corrigeant une inégalité de traitement entre les titulaires de ces pensions. Alors que le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis a été commémoré en 2017, l'année 2018 marquera la fin du cycle mémoriel consacré au centenaire de la Grande Guerre. Le budget de la politique mémoire a été largement augmenté. augmenté. À cet égard, je tiens à saluer l'initiative du Gouvernement d'accroître de 5,3 millions d'euros le budget consacré aux commémorations de la Grande Guerre, afin de permettre aux opérateurs d'organiser toutes les cérémonies prévues à ce titre. titre. Le représentant de la Meuse que je suis y est très sensible, et je pense que les élus de mon territoire, au regard de l'historique bataille de Verdun, le seront aussi. Par ailleurs, je me réjouis de l'affectation de 11,2 millions d'euros à l'entretien, à la rénovation et à la valorisation de nos monuments et lieux de mémoire. La mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » joue aujourd'hui un rôle essentiel, permettant la réconciliation de différentes générations autour de notre bien commun : la Nation et son histoire. Ce budget est marqué par le souci de la transmission de la mémoire, notamment à la jeunesse. Elle est, à mon sens, primordiale. Bien menée, elle permet aux jeunes de s'approprier leur histoire, tout en associant les différentes générations de Français autour de la Nation. Une réflexion doit être menée afin de rendre le devoir de mémoire plus audible pour les jeunes générations. Il faut donner une nouvelle dimension, une nouvelle dynamique aux activités destinées à pérenniser le devoir de mémoire. La direction du patrimoine, de la mémoire et des archives me semble être la structure la plus à même de remplir cette mission. Pour terminer, je souhaiterais m'attarder quelques instants sur les perspectives d'avenir du monde combattant contemporain. Celui-ci regroupe les Français et les personnels des anciennes colonies ayant participé à la Seconde Guerre mondiale, aux guerres d'Indochine d'Afrique du Nord, mais également aux opérations extérieures. Il est également composé des victimes de guerre et du terrorisme. Aujourd'hui, la génération des opérations extérieures n'adhère que trop faiblement au monde combattant. À moyen terme, il serait important que ces combattants intègrent les associations patriotiques et le monde combattant, afin que les actions de reconnaissance ne se limitent pas aux acquis des générations précédentes. En effet, les participants aux opérations extérieures, les victimes de guerre et du terrorisme sont les représentants du monde combattant contemporain. Pour préparer l'avenir, des mesures doivent être prises. Je pense notamment aux soldats engagés en Afrique du Nord entre le 2 juillet 1962 et le 1 juillet 1964 pour assurer le transfert de nos installations.

et le système d'attribution au titre des opérations extérieures n'a été créé que postérieurement. Il serait souhaitable qu'ils puissent obtenir la carte du combattant et la croix du combattant, au même titre que les forces engagées dans les OPEX, et qu'ils puissent ainsi bénéficier de la retraite du combattant, sans effet rétroactif- je ne demande pas l'impossible Madame la secrétaire d'État, il est nécessaire de mener une réflexion approfondie sur le sujet, afin de combler le vide juridique sur ce dossier et d'attribuer à ces hommes la reconnaissance qu'ils méritent. Pour conclure, Verdun étant Verdun étant le symbole de la Première Guerre mondiale, l'inscription de ce champ de bataille au patrimoine de l'UNESCO serait à mon sens le plus parfait des aboutissements du centenaire de cette guerre. Le groupe du RDSE soutient l'action du Gouvernement et votera en faveur de ce budget.

mémoire et liens avec la Nation » du quinquennat tient la double promesse du Gouvernement de maîtriser les finances publiques tout en renforçant les dispositifs et les projets de cette mission, avec un budget de 2,46 milliards d'euros. Des trois programmes qui composent la mission, le troisième, le programme 158, relève de la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et rassemble trois dispositifs en faveur des victimes de la Seconde Guerre mondiale ou de leurs ayants cause. Son budget de 100,8 millions d'euros, inchangé par rapport 46,4 millions d'euros, à l'indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes spoliées par les législations antisémites de l'Occupation et, pour 54,3 millions d'euros, à l'indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Le programme 169, quant à lui, concentre la quasi-totalité des crédits de la mission, avec 2,32 milliards La baisse de 3,3 % en autorisations d'engagement pour 2018 est le reflet d'une diminution progressive du nombre des bénéficiaires des différents dispositifs, malgré l'arrivée de la quatrième génération du feu, avec les combattants des opérations extérieures. Pour autant, plusieurs des prestations ont été ou vont être revalorisées au profit des anciens combattants. Tout d'abord, la hausse de deux points de la retraite du combattant est entrée en vigueur le 1 septembre 2017. En 2018, pour porter

Le calcul se fera désormais sur la base du grade, pour un coût de 6 millions d'euros. Enfin, une mesure spécifique du budget pour 2018 revalorise de 100 euros les deux allocations versées aux anciens membres des formations supplétives, allocations qui progresseront respectivement de 4,2 % et 5,5 %. Cette mesure est un renforcement bienvenu de la reconnaissance de la Nation à l'égard des harkis et de leurs familles. Le programme 167, « Liens entre la Nation et son armée », rassemble les crédits consacrés à la mémoire combattante et ceux qui La forte progression des crédits de ce programme correspond à la dernière année du cycle mémoriel du centenaire de la Première Guerre mondiale, notamment la commémoration du 11 Novembre, qui donnera lieu à une cérémonie internationale 8 millions d'euros seront versés à la Mission du centenaire. De plus, une enveloppe de 12,4 millions d'euros sera consacrée à la valorisation du patrimoine de mémoire, des sépultures et hauts lieux de la mémoire nationale. Le développement du tourisme de mémoire, qui connaît un regain avec le centenaire, doit bien entendu être poursuivi, notamment avec l'implication des collectivités locales. L'année 2018 sera également une année importante pour la stratégie ministérielle globale en direction des jeunes. La direction du service national et de la jeunesse est désormais chargée de coordonner l'ensemble des actions du ministère liées à la politique du service national, à l'insertion et à la lutte contre les exclusions. Elle disposera d'un budget de 14,6 millions d'euros. Chaque année, 800 000 jeunes participent à la journée défense et citoyenneté, ou JDC, un jalon essentiel de leur parcours citoyen. La JDC leur apporte une information sur les enjeux de la sécurité nationale, mais représente également une opportunité de prolonger cette prise de conscience par diverses formes d'engagement, de la réserve opérationnelle au service civique. Fidèle à sa mission de cohésion sociale, la JDC permet aussi de repérer et d'apporter un soutien ciblé aux jeunes décrocheurs, qui peuvent se voir proposer de rejoindre l'EPIDE, ou le service militaire volontaire, dont les premiers résultats prometteurs justifient pleinement la reconduction jusqu'au 31 décembre 2018. Pour approfondir et renforcer encore le lien entre les jeunes Français et les armées, le Président de la République souhaite la création d'un service national universel. La réflexion en cours permettra d'associer toutes les parties prenantes de la communauté nationale, tant il est vrai que le ministre des armées ne peut, seul, porter ce projet structurant. Madame la secrétaire d'État, les crédits de cette mission montrent que 2018 sera une année charnière, avec de nombreux projets en cours que vous nous avez exposés avec beaucoup de clarté lors de votre audition par la commission des affaires sociales. Je vous remercie sincèrement de la qualité de votre écoute. C'est là une heureuse marque de fabrique de l'action conduite par le Gouvernement et sa majorité, sous l'impulsion du chef de l'État. Le groupe La République En Marche votera ces crédits, bien entendu, et vous accompagnera sur le chemin des réformes à venir,

qui visent à spéculer sur la baisse démographique, et donc sur la mort de ceux qui ont combattu pour la France, de ces femmes et de ces hommes à qui nous devons beaucoup. Nous ne pouvons parler des anciens combattants sans regretter la suppression du secrétariat d'État qui Cette décision en dit long sur la place qu'occupent ces femmes et ces hommes dans l'esprit du Gouvernement et du Président de la République. Aujourd'hui, la réalité est là : les anciens combattants ne sont plus qu'un dossier parmi d'autres au ministère des armées, et l'on continue de faire des économies sur le dos de personnes qui ont tant donné La baisse constante du budget depuis plus de dix ans ne permet pas de répondre aux demandes récurrentes et au droit à réparation du monde combattant. Les iniquités et les frustrations persistent, mais nous considérons, au groupe communiste républicain citoyen et écologiste, qu'elles peuvent être résolues par des chiffrages actualisés

Évidemment, nous pouvons nous féliciter de la revalorisation de la pension versée aux harkis, forces supplétives de l'armée française lors de la guerre d'Algérie. Cette revalorisation ne peut toutefois cacher les manques de ce budget. des injustices entre les différentes générations d'anciens combattants. Pourtant, comme l'a très bien souligné mon collègue André Chassaigne à l'Assemblée nationale, « celui qui a combattu a combattu, celui qui est mort est mort, et l'on ne doit pas faire de différence ».

pour la France, sur la revalorisation de la pension de base des conjoints survivants des grands invalides de guerre, ou encore sur la demande des harkis de souche européenne de bénéficier de l'allocation de reconnaissance, en dépit du refus réitéré opposé par le Conseil constitutionnel

Pouvons-nous aussi évoquer le fait que le statut d'ancien combattant ne soit toujours pas accordé aux militaires français déployés en Algérie entre 1962 et 1964 ? Ceux qui ont perdu la vie pendant cette période ont droit à l'appellation « mort pour la France », les autres à un titre de reconnaissance de la Nation, et si l'État français accorde

même peloton et y ont effectué, ensemble, les mêmes missions, les mêmes jours, aux mêmes horaires ? L'excuse selon laquelle la guerre a pris fin le 2 juillet 1962 n'est pas justifiable.

j'aurai un mot pour les veuves, des femmes qui ont eu la douleur, mais apparemment aussi le tort de perdre leur mari avant que ce dernier atteigne l'âge de 74 ans, puisqu'elles sont privées de la demi-part fiscale ... Sommes-nous conscients que cette décision est une double peine ? aux veuves de grands invalides qui, du fait de l'état de dépendance de leur époux, se sont consacrées à lui en permanence au détriment d'une carrière professionnelle et qui, au décès de ce dernier, n'ont pu bénéficier que d'une très modeste pension de réversion. Nous devons agir à leur égard. Vous le savez, madame la secrétaire d'État, la liste des inquiétudes est encore longue ... Face à cette situation, l'État a le devoir de ne pas se défiler, car il est de son ressort qu'il n'y ait aucun oublié de la République. Je terminerai mon intervention en disant que le présent projet de loi de finances va creuser davantage les inégalités, car la baisse du budget des anciens combattants accompagne aussi la baisse des APL et la hausse brutale de la CSG,

ce débat est un moment fort de nos discussions sur le projet de loi de finances et présente, en somme, des enjeux majeurs. En effet, il constitue une étape importante qui traduit l'engagement de la France vis-à-vis de son passé, mais aussi, dans un certain sens, de son avenir. Car, au fond, c'est bien de cela qu'il est question aujourd'hui : la reconnaissance de la Nation pour ses combattants, toutes générations confondues, et la transmission de ce témoin de l'Histoire aux générations futures. Comme le dit si bien cette formule faisant référence à Simone Veil, à qui je veux rendre hommage : « Transmettre la mémoire de l'Histoire, c'est apprendre à se forger un esprit critique et une conscience ». Alors, tout d'abord, je ne vous cacherai pas notre déception concernant ce texte. La volonté est là, mais les moyens déployés demeurent en deçà des objectifs fixés. Année après année, majorité après majorité, les gouvernements successifs s'entêtent dans la baisse des crédits alloués à cette mission, pourtant si fondamentale. Ainsi, le budget pour 2018 s'établit à 2,46 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une baisse de 3,1 %. Si l'on en croit la loi de programmation des finances publiques, la baisse cumulée sera de 11,4 % en 2020. Cette situation est inacceptable pour nos combattants d'hier et d'aujourd'hui, leurs conjoints et leurs descendants. Ces soldats ont participé à l'effort de guerre en payant parfois un lourd tribut. Ils méritent donc plus de considération et ne doivent pas être une simple variable d'ajustement des comptes publics. Alors, si cette baisse dégage des économies pour l'État, elle n'en est pas moins ressentie comme un renoncement, voire une résignation. C'est notamment le cas pour le programme 169, destiné à la reconnaissance et à la réparation en faveur du monde combattant. Ses crédits diminuent eux aussi de 3,4 %. Cette évolution peut s'expliquer par la réduction du nombre de bénéficiaires. Nous entendons et comprenons cet argument. Toutefois, la dynamique démographique ne justifie pas tout. En effet, les défis à relever sont multiples, et les demandes nombreuses. Conscients de ce changement, nous vous demandons, non pas d'augmenter ces crédits, mais de les maintenir à leur niveau actuel. Pour ainsi dire, nous regrettons l'absence de mesures fortes. Comme l'indique le rapporteur pour avis dans son rapport, ce budget « ne corrige en aucun cas les insuffisances du droit à réparation et les inégalités que son application engendre. » Nous aurions aimé que des solutions soient apportées aux pertes de pouvoir d'achat. Si l'extension en année pleine de la revalorisation de la retraite du combattant s'inscrit dans le bon sens- nous tenons à le souligner -, les mesures demeurent encore trop insuffisantes. Par ailleurs, je veux attirer votre attention sur deux sujets importants, relayés par de nombreuses associations. Le premier concerne l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation pour les personnels engagés dans l'opération Sentinelle. Ces femmes et ces hommes exercent leur devoir dans des conditions difficiles, parfois même déplorables : temps de repos, hébergement, logistique, problèmes de matériel, etc. Nous ne pouvons pas rester insensibles à cette situation. Ces héros de la République risquent chaque jour leur vie et sont régulièrement la cible de fanatiques. Par conséquent, il serait souhaitable de les considérer comme des combattants à part entière et, de manière générale, de revoir ce dispositif pour les missions intérieures. Le second sujet concerne l'octroi de la carte du combattant au titre d'une OPEX pour les opérations de sécurité conduites sur le territoire algérien après le 2 juillet 1962, en application des accords d'Évian. Il s'agit non pas de travestir l'Histoire, mais de rétablir des faits. Une proposition de loi a d'ailleurs été déposée en ce sens à l'Assemblée nationale, en 2012, par ... M. Gérald Darmanin. Nous comptons donc sur le Gouvernement pour pallier cette injustice. N'attendons pas qu'il n'y ait plus d'anciens combattants pour prendre en considération ce qu'ils demandent depuis tant d'années Aussi, nous saluons le choix fait d'augmenter les crédits pour la politique de mémoire. Les différentes commémorations prévues, notamment celles qui sont liées à la Première Guerre mondiale, témoignent de cette volonté forte de nos institutions de renforcer les liens entre les citoyens et les armées. Nous nous en réjouissons. La quatrième génération du feu sera également mise à l'honneur, notamment lors du quarantième anniversaire de la force intérimaire des Nations unies au Liban. L'actualité au Proche-Orient nous rappelle l'importance de l'amitié franco-libanaise, mais aussi le rôle déterminant de notre pays dans le concert des nations. ailleurs, nous rejoignons l'avis du rapporteur spécial sur l'indemnisation des victimes de persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle mérite en effet de « recevoir un nouvel élan Concernant la journée défense et citoyenneté, il paraît nécessaire de la recentrer sur sa vocation première : l'esprit de défense. L'impact financier du service national universel changera considérablement les choses. C'est une mesure attendue, qui, j'en suis sûre, fera l'objet d'un débat parlementaire à la fois riche et constructif. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'intervenir sur ce sujet dès le mois de janvier 2018. Pour terminer, nous soutenons le Gouvernement s'agissant des deux articles rattachés. La revalorisation de 100 euros des deux allocations versées aux anciens membres des formations supplétives et l'harmonisation des pensions militaires d'invalidité versées aux ayants droit des militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 constituent une évolution positive. À ce propos, le temps est venu d'ouvrir un débat apaisé, de mettre enfin des mots sur une période difficile, complexe et si douloureuse pour nos compatriotes harkis. Ils ont connu les pires atrocités ; nous aspirons pour eux à plus de justice et de reconnaissance.

Surtout, derrière les chiffres et les discussions budgétaires se cachent avant tout des noms, des visages et des vies consacrées. Ne les oublions pas ! La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, messieurs les présidents de commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, honorer nos combattants, honorer leur engagement, honorer leur mémoire, nous le faisons lors des différentes manifestations patriotiques et des remises de décorations. Mais nous ne devons surtout pas oublier de le faire aussi chaque année à l'occasion de l'examen du budget des anciens combattants, pour respecter le droit à la reconnaissance et à la réparation. Madame la secrétaire d'État, les budgets des anciens combattants se suivent et se ressemblent. Ils sont en baisse régulière. La diminution pour 2018, de l'ordre de 3 %, est une nouvelle fois justifiée par la baisse naturelle des bénéficiaires, mais surtout par la rigueur budgétaire. Nos anciens combattants doivent-ils subir et être l'otage de la rigueur budgétaire ? Personnellement, je ne le pense pas. Il est vrai que, une fois de plus, vous n'avez pu obtenir de Bercy le bénéfice d'un budget constant. Si tel avait été le cas, cela vous aurait permis de prendre en compte les principales revendications maintes fois soulevées depuis plusieurs années par le monde des anciens combattants. Dans ce contexte budgétaire difficile, vous avez tenu à maintenir l'ensemble des dispositifs de reconnaissance et de réparation. Vous avez également tenu à honorer les engagements pris par le précédent gouvernement en finançant, en année pleine, l'augmentation de la retraite décidée l'année dernière. Vous avez aussi tenu à prévoir dans le budget les crédits nécessaires pour marquer les événements qui vont clore le cycle mémoriel du centenaire. Vous avez enfin Vous avez enfin tenu à mettre en oeuvre plusieurs mesures nouvelles : l'harmonisation des pensions de réversion des conjoints de militaires, la revalorisation des droits des anciens membres des forces supplétives, l'amélioration des dispositifs de réparation en faveur des harkis. Malgré ces mesures appréciées du monde des

entendu leurs requêtes maintes fois réitérées depuis plusieurs décennies. C'est vrai ! Ils demandent depuis longtemps que la valeur du point servant de calcul à plusieurs dispositifs, et déterminée selon le rapport constant, puisse être actualisée. Ils demandent que le bénéfice de la campagne double soit attribué en fonction du temps passé sur un territoire de guerre, et non plus des actes de feu. Ils demandent le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves dont le mari est décédé avant 74 ans.

Madame la présidente, messieurs les présidents de commission, monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer le travail réalisé par M. le rapporteur spécial pour avis sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». J'ai une amicale pensée pour Bruno Gilles, mon collègue des Bouches-du-Rhône actuellement hospitalisé, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement et que nous espérons retrouver très vite dans cet hémicycle. En ma qualité de membre du groupe d'études des sénateurs anciens combattants et de la mémoire combattante, j'avais exprimé dès le mois de mai le malaise de bon nombre d'associations qui avaient fait part, dans nos dans nos territoires, de leurs interrogations en l'absence d'un ministère de plein droit qui leur soit dédié. Aussi, madame la secrétaire d'État, si votre nomination auprès du ministre des armées est une bonne chose, des signes de reconnaissance doivent être envoyés par le Gouvernement qui sont transmis par le budget 2018 sont en demi-teinte. C'est d'autant plus regrettable que l'année 2018 viendra clore le cycle mémoriel consacré à la Grande Guerre. Et vous savez combien les symboles sont importants en matière de lien entre la Nation et son armée à l'heure où la République doit promouvoir les valeurs de la citoyenneté. Il y a beaucoup à dire sur un budget en perpétuelle diminution- la baisse est de 3 % par rapport à 2017 -, dans lequel, malheureusement, les injustices perdurent et les prestations à caractère universel sont dévalorisées au profit d'avantages plus sélectifs. Bien sûr, le nombre de bénéficiaires est à la baisse. Pour autant, de nombreux points restent encore en suspens : la revalorisation significative de la retraite, la demi-part part fiscale pour les veuves ayant perdu leur conjoint avant 74 ans, l'octroi de la carte du combattant aux militaires déployés en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1 juillet 1964, la reconnaissance de la Nation envers les pupilles, la situation des conjoints survivants des grands invalides, les supplétifs de statut de droit commun. Je tiens à souligner le travail effectué sur les territoires par les associations, ainsi que par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui tisse des liens et des passerelles. Dans un contexte qui s'est beaucoup modifié ces dernières années, je m'interroge toutefois sur notre organisation actuelle. En effet, avec la prise en charge, d'une part, des opérations extérieures et de la quatrième génération du feu et, d'autre part, des victimes d'actes de terrorisme, les missions et les besoins ont considérablement évolué. Pour m'être rendue, voilà quelques jours, au 4 régiment de chasseurs de Gap à l'occasion de la dissolution du Groupement tactique blindé Edelweiss, je sais combien certaines situations sont préoccupantes et combien elles nécessitent attention, bienveillance et accompagnement. C'est pourquoi nous devons veiller à prendre en compte la situation des blessés, qu'ils le soient physiquement ou psychologiquement. Ces hommes et ces femmes doivent être accompagnés sur le chemin de la guérison, mais aussi sur celui de la réinsertion professionnelle. Un effort doit également être fait en direction des aidants, notamment des grands invalides de guerre. J'espère que nos discussions nous permettront d'avancer sur tous ces sujets, même si nous savons que certains points font actuellement l'objet de rapports qui devront être étudiés ultérieurement. La parole

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs,

Mais le monde combattant est bien sûr prioritaire dans les missions qui m'ont été confiées par Florence Parly et par le Premier ministre. J'ai bien entendu

plusieurs dizaines d'années. Vous voudrez bien me faire grâce du fait que je ne peux pas régler tous ces problèmes en un

est à M. Philippe Mouiller. Au sein de la troisième génération du feu, qui a servi en Algérie, une dernière inégalité persiste dans l'attribution de la carte du combattant. Depuis 2004, celle-ci est attribuée à tous les hommes qui y ont servi quatre mois avant l'indépendance, c'est-à-dire le 2 juillet 1962. Depuis 2014, tous les soldats qui ont servi quatre mois sur ce territoire, dès lors que leur séjour avait commencé avant cette date, peuvent la recevoir- c'est ce qu'on appelle la carte « à cheval Cela ne prend pas en compte la situation des militaires qui, en application des accords d'Évian, ont été affectés dans ce pays nouvellement indépendant jusqu'en 1964, dont l'effectif total est estimé à plus de 150 000 hommes.

Pour le Gouvernement, il représenterait plus de 100 millions d'euros, mais ce calcul est basé sur l'hypothèse que l'ensemble des soldats concernés n'en bénéficient pas aujourd'hui et la percevront dès l'an prochain. Or un nombre important de ces hommes avait déjà servi en Algérie durant la guerre et touche la retraite du combattant à ce titre. Il est plus raisonnable d'estimer qu'environ 25 000 personnes seraient concernées, soit le nombre de titres de reconnaissance de la Nation décernés pour les services en Algérie entre 1962 et 1964- environ 36 000 duquel est soustrait le nombre de cartes « à cheval » attribuées depuis 2014- 11 000. Le coût serait donc d'environ 18 millions d'euros par an, ce que le déclin démographique des anciens combattants permet de financer à budget constant. Par ailleurs, il n'est pas question en l'occurrence de rouvrir le débat sur la guerre d'Algérie et ses bornes temporelles. Le maintien de forces françaises sur ce territoire indépendant après le 2 juillet 1962 s'apparente plutôt à une opération extérieure. depuis 2015, les anciens combattants des OPEX peuvent bénéficier de la carte du combattant après quatre mois de présence sur un théâtre d'opérations. Ces OPEX ne sont pas toutes postérieures à la guerre d'Algérie : dans la liste, fixée par arrêté, on compte par exemple Madagascar entre mars 1947 et octobre 1949. l'intervention du législateur ne serait donc même pas nécessaire, si le Gouvernement prenait ses responsabilités. Il lui suffirait en effet de modifier cet arrêté. En raison des règles propres à la recevabilité des amendements au projet de loi de finances, cet amendement prévoit le transfert de 18 millions d'euros de l'action n° 02 vers l'action n° 01. L'amendement

de campagne : en effet, le 25 avril 2017, il s'est adressé aux associations du monde combattant, en se déclarant « favorable à l'attribution de la carte du combattant aux militaires déployés en Algérie entre le 3 juillet 1962

Nous sommes au lendemain de la journée commémorative de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc et le Président de la République est à Alger aujourd'hui même. Nous sommes donc à un moment où la question de l'attribution de la carte du combattant aux soldats français engagés- appelés, pour beaucoup d'entre eux -en Algérie de 1962 à 1964 doit être posée. Les plus jeunes de ces soldats ont aujourd'hui 73 ans.

Pour la réconciliation franco-algérienne, la reconnaissance de l'engagement des soldats français en Algérie

Le pragmatisme est évidemment important, surtout en période de crise budgétaire. Néanmoins, si notre politique ne fait pas sens, je ne vois plus la signification réelle du mot « politique ». Opposer la rigueur budgétaire à ces anciens combattants serait indigne.

Lorsqu'il s'est agi, il y a quelques jours, de voter la hausse de la CSG qui risquait de frapper nos anciens, nous avons refusé, au Sénat, et nous avons eu raison. Aujourd'hui, nous devons protéger et honorer nos anciens combattants.

certains ont servi avant 1962 et d'autres après. S'ils ont parfois des médailles, ils n'ont pas la même carte du combattant. J'aimerais leur dire que, aujourd'hui,

demandes. Je souhaite que chacun reconnaisse que le travail n'a pas été fait auparavant

Mme Corinne Féret. Cet amendement concerne la situation des anciens combattants qui, contrairement à leurs veuves, ne peuvent bénéficier d'une aide complémentaire,

d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Un consensus existe au sein de la représentation nationale, mais nous devons maintenant le rendre effectif. En l'an 2000, le Gouvernement a en effet reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes pendant la guerre de 1939-1945. Dès la fin 2001, le Gouvernement a été sollicité pour que d'autres orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie puissent bénéficier des mêmes indemnisations que les victimes de la Shoah. À l'époque, le secrétariat d'État chargé des anciens combattants avait organisé la mise en place d'une commission pour répondre à cette nouvelle demande, ce qui avait abouti à la publication du décret de 2004, lequel s'adresse aux orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Une troisième catégorie de pupilles de la Nation, souvent déboutée dans le cadre des décrets de juillet 2000 et de juillet 2004, sollicite la reconnaissance de la part de l'État, celle dont les parents résistants sont morts les armes à la main et sont reconnus par la mention marginale portée sur les registres d'état civil « Mort pour la France ». Il s'agit, à travers cet amendement, de permettre à toutes et tous cette reconnaissance de pupille de la Nation.

nature du dispositif, lequel a été mis en oeuvre pour des situations très particulières d'orphelins de parents morts en déportation, ainsi que d'orphelins de parents parents qui auraient subi la barbarie nazie dans les camps de déportation, les camps de la mort. La cible est tout à fait

ramène en arrière, au moment de la commission Mattéoli. La question était de savoir si nous reconnaissions ou non la défaillance de l'État français. Quelle est sa responsabilité vis-à-vis des crimes de la barbarie nazie ?

souvent le père -morts pour la France au titre de leur mission de soldat et dans le cadre de la défense du territoire et du pays, lors d'une guerre,

dans les formations supplétives et ont connu exactement les mêmes conditions de vie et d'engagement que leurs camarades musulmans. Pourtant, plus de 55 ans après les faits, l'allocation de reconnaissance leur est toujours refusée, bien qu'ils aient bénéficié, entre 2011 et 2013, de décisions de justice en leur faveur.

Malgré des décisions favorables prises à leur égard par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, leur situation n'est toujours pas réglée. Du fait de leur âge avancé- ils ont en moyenne 80 ans -, les supplétifs de statut civil de droit commun sont de santé précaire.

seuls 70 supplétifs de statut civil de droit commun pourront prétendre à l'allocation de reconnaissance. La rente annuelle

anciens supplétifs en tenant compte de la situation spécifique de ceux dont le statut civil, en Algérie, relevait du droit commun et non du droit local

débat n'a que trop duré au regard de l'âge de ces anciens combattants, dont l'état de santé se dégrade. Tous les élus ont été sollicités à ce sujet, Il est temps, à mon avis, de clôturer ce chapitre et, surtout, de refermer les plaies incompatibles avec la volonté d'apaisement nécessaire à toute politique de mémoire. La parole est à Mme Corinne

disparaître. La très grande majorité des harkis relevaient du statut civil de droit local. Toutefois, des pieds-noirs, de statut civil de droit commun, se sont engagés à leurs côtés dans les différentes formations supplétives. Le législateur leur a toujours refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance. Une décision du Conseil constitutionnel de 2011 leur a donné satisfaction, mais l'administration n'a pas accédé à leurs demandes et une loi de 2013 les a de nouveau exclus du dispositif. Environ 70 personnes seraient concernées,

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits, modifiés.

du rapport constant, sur l'augmentation du point d'indice pour les pensions militaires et la retraite du combattant et sur les conditions d'octroi de la demi-part supplémentaire pour les veuves de titulaires de la carte du combattant, afin que nous puissions disposer de l'ensemble de ces éléments. L'amendement

Désormais, la très grande majorité des anciens combattants, notamment ceux d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, ainsi que 85 % des bénéficiaires de la retraite du combattant sont effectivement âgés de plus de 75 ans. Néanmoins, il demeure une injustice majeure entre les veuves d'anciens combattants. En effet, celles dont le mari est décédé tôt, avant 74 ans, sans avoir donc pu bénéficier de cette demi-part, ne peuvent dès lors en bénéficier. Cela concerne 40 % des veuves d'anciens combattants.